La séance est ouverte. Le compte rendu analytique, la précédente séance a été distribué il y a pas d'observation, le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle les. Ponce Ponce à des questions orales. La parole est à madame Nadia Sollogoub. Je vous en prie, chers collègues. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le cas de certaines petites petites communes rurales qui sont contributrices au Fonds national de garantie individuelle des ressources. Le FN GIR de dont le montant depuis 2014 et figé alors que les ressources de ces mêmes communes par ailleurs évolue et en général de façon plutôt négative, alors j'aimerais savoir et j'avais porté des amendements en ce sens-ci serait envisagé sa chambre de bonne logique que en deux ça d'un certain seuil de population de pouvoir et exonérer les plus petites communes de contribution au FN GIR, je vous remercie. Madame la Ministre. Merci monsieur le le président, madame la sénatrice. Bon alors je je peux d'abord vous indiquez vous le savez que le dispositif en vigueur a permis d'assurer une stricte neutralité financière pour chaque collectivité locale. L'article 78 de la loi de finances pour 2010, qui a prévu un mécanisme pérenne destinée à assurer cette neutralité. Se compose comme vous le savez d'une dotation de. Compensation de la réforme de la taxe professionnelle financée par l'État et du FN GIR dont vous nous parlez dans votre question. À un prélèvement ou un renversement au titre du FNJ re-calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après la réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010 au terme d'une opération à caractère national. Depuis 2012, les montants prélevés ou. Reversés au titre du FNE GIR son fixe en euros constants, ce qui permet d'éviter une instabilité des compensations. Les montants de prélèvement ou des reversements au titre du FNE GIR sont désormais figées cette fixité offrent une stabilité aux collectivités territoriales est n'est pas structurellement pénalisante pour les contributeurs qui ont connu depuis 2010, un dynamisme de leur fiscalité économique local leur contribution au FN GIR n'a pas augmenté, tandis que leurs ressources fiscales ont augmenté. l'objectif du législateur et tente de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps la réactualisation, année après année des prélèvements alimentant le FNJ. Leur réfaction dégressives ne paraît guère envisageable toutefois le gouvernement est pleinement conscient des difficultés liées à la fixité du FN pour les communes contributrices notamment rurales dont vous parlez, madame la sénatrice, qui sont confrontés au départ d'une ou plusieurs entreprises de leur territoire. Des mesures ont été prises pour compenser les pertes exceptionnelles de base de contribution économique territoriale. D'une part l'article 79 de la loi de finances pour 2021 a créé un prélèvement sur recettes de l'État. Prévoyant que l'État verse. Annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au Fonds national de garantie individuelle des ressources pour les communes qui acquitte un prélèvement au titre du FNE GIR représentant plus de 2% de leur recettes réelles de fond. Même la ministre et le temps est largement dépassé les notes qu'on vous fait il faudrait bien n'est pas trop merci je le dirai à Bercy. Voilà, merci. Madame ce logo. Oui mais. Merci madame la mise. J'entends bien en effet que cette note a été préparée par Bercy et mais malgré tout, si vous voulez, concrètement, moi je vous donne le cas de la commune de base dans la Nièvre. 290 habitants y contribue au fait dire pour 50.000 euros alors la fixité en effet pour eux, le seul problème, c'est pas la fixité c'est c'est le montant et quelque part, ça semble complètement déraisonnable. Alors j'avais porté des amendements au projet de loi de finances, on m'avait répondu qu'il peut y avoir des toutes petites communes. Malgré tout, avec un fort potentiel fiscal des Mais concrètement, même s'il y a sur cette commune des habitants qui qui sont relativement aisée riche ça apporte absolument pas d'argent dans la caisse de de la de la municipalité qui doit faire face à la réfection des routes et à la réfection du du toit de l'église ça change rien du tout à son budget et non seulement ça mais même si on imaginait. Un cas extraordinaire qui a un millionnaire, sur la commune de base l'. On pourrait pas augmenter la fiscalité pour l'ensemble des habitants, parce que sous prétexte qu'il y en a un qui est beaucoup plus riche que les autres et d'autant plus que depuis la réforme de la taxe d'habitation, ça rapporterait encore. Rien du tout. Le levier fiscal quelque part n'existe plus. Donc en même temps qu'on a réformer la taxe d'habitation. taxe d'habitation. Il aurait fallu. Les toutes petites communes qui peuvent plus disposer du levier fiscal, dans leur collectivité et qui se retrouvent avec des Budgets avec des des aberrations quelque part donc voilà je reformule ma demande et puis je la reformule. Chaque année. Nous avons confiance. La parole est maintenant monsieur Daniel Salmon. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre après 2 années d'expérimentation du menu végétarien dans la restauration collective mise en place par la loi climat et résilience expérimenté dans plus de 200 communes, un consensus émergeait sur les bienfaits de ce menu équilibré pour la bonne santé des enfants et vertueux pour l'environnement. Pourtant un nouvel arrêté ministériel en cours d'écriture pourrait imposer une quantité minimale de viande et de poisson dans les cantines. Le résultat de la contre-offensive de l'industrie agroalimentaire qui pourrait rendre impossible l'alternative végétarienne pour la restauration scolaire. Or les bénéfices des repas végétariens sont multiples, d'abord pour la santé. Réduire notre consommation de viande permet de réduire les risques de maladies chroniques d'origine nutritionnelle comme l'obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires encore les cancers lancé ça a confirmé qu'un menu végétarien équilibré apporte la quantité de protéines nécessaires à la santé. Ensuite les économies réalisées grâce aux menus végétariens serve à introduire plus de viande bio et local. 20% des cantines sans menus végétariens proposent de la viande bio, local contre 50% des cantines avec un menu végétarien quotidien un cercle vertueux bénéficiant ainsi à toutes les parties prenantes. Le menu végétarien est aussi un modèle d'inclusion selon le défenseur des droits, ils constituent une alternative. De frein éthique religieux ou sociaux. Il était également bénéfique bien sûr pour le climat, l'alimentation représente 24% de l'empreinte carbone des ménages français chaque repas végétariens évite l'émission de 1,5 kilos de carbone en moyenne, soit environ 10 kilomètres en voiture, il est indispensable d'adapter notre système alimentaire aux enjeux climatiques et aux limites planétaires Madame la Ministre plutôt que de mettre un terme à une expérimentation qui a fait ses preuves. Pérennisons là. Laissons famille le choix de leur alimentation pouvez-vous vous engager à l'occasion du nouvel arrêté cantine à permettre à toutes les cantines du 1er et du second degré de servir une option végétarienne sur une base quotidienne. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur. Le rapport relatif à l'expérimentation de l'option végétarienne quotidienne pour les collectivités volontaires est en cours d'élaboration. Sur la base des travaux d'une mission inter. Inter inspection associant celle de l'agriculture et de l'environnement. Seuls 49 collectivités ont souhaité s'inscrire dans ce cadre de dans le cadre de cette expérimentation et partager cette expérience sur les 200. Que vous Que vous avez cité des entretiens qualitatifs complémentaires ont ainsi dû être organisé par la mission. Depuis 2012, il est obligatoire de servir sur 20 repas successifs du poisson lors de 4 repas de la viande rouge non hachée lors de 4 repas en cas de choix multiples. Il est donc possible de servir une option végétarienne quotidienne dès lors que l'avion de la viande et du poisson sont servis dans les options non végétarienne de même certaines collectivités ont mis en place une option végétarienne. Surréservation quelques jours à l'avance ce qui s'apparente bien à un choix multiple. En revanche le cadre existant depuis 10 ans ne permet pas une inscription à une option végétarienne à l'année ou au trimestre. Car de fait les Elham inscrit à cette option n'auront pas la possibilité de manière certaine de consommer de la viande ni du poisson pendant toute une année ou un trimestre cette interprétation a d'ailleurs été confirmée par le tribunal administratif de Lyon qui a estimé le 23 mars 23 que la décision de la mairie de Lyon d'instaurer des menus sans viande du 22 février au 2 avril était contraire au respect de la qualité nutritionnelle des repas. rappelle que la recommandation de la du Haut comité de santé publique pour les enfants sont en effet de consommer du poisson 2 fois par semaine, de la viande de volaille et tous les jours sans qu'il soit nécessaire d'en consommer à chaque repas. Merci monsieur seulement vous avez 4 secondes. Mais allez. Ça va être court. Non, mais clairement il va falloir faire évoluer les pratiques et les mauvais, régimes alimentaires, c'est écrit dans tous les rapports, les rapports du GIEC le montre sans évolution de notre régime alimentaire on n'arrivera pas atteindre les trajectoires pour réduire les gaz à émission de serre. Il merci Madame Espagnac. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre cette question. S'adresser à monsieur Berville, le ministre de la mer et en charge des des pêcheurs Madame la Ministre. Le 29 mars dernier, les marins-pêcheurs ont décidé de bloquer le port de Bayonne pour alerter sur la leur situation et leurs inquiétudes quant à la à venir, venant d'Arcachon ou de Cap-Breton il. A raison. A raison. La décision du Conseil d'État du 20 mars dernier qui ordonne au gouvernement de fermer des zones de pêche dans le Golfe de Gascogne pour une durée totale qui pourrait être de quatre mois dans un de lits de six mois, si chacun ici je le pense, partage l'objectif de d'effort de la biodiversité et tout particulièrement ne doit pas s'il ne doit sa pas se faire en aucun cas pardon au détriment de nos pêcheurs. Cependant, après un plan de sortie de flotte dégradant les capacités de pêche la décision. Suite de la Commission européenne d'interdire le chalutage dans les aires marines protégées d'ici 2030. Voici le Conseil d'État qui charge encore la barque nous marins-pêcheurs qui était déjà dans une situation compliquée et risque de voir leur chiffre d'affaires baisser jusqu'à 50% si durant un tiers de l'année des zones de pêche leur sont supprimés ce sont près de 3000 marins et familles qui risque d'être affectés par cette décision qui fait courir un risque majeur pour la filière de la pêche secteurs importants de notre économie, ces pêcheurs qui exercent leur métier avec passion un métier aux conditions difficiles ne peuvent entendre que l'État leur supprime une partie de leur travail. Il est urgent de trouver des solutions qui à la fois protégeront les dauphins et les pêcheurs et qui leur permettront à nouveau de retourner au large et de larguer les amarres plutôt que de jeter l'éponge. Ces derniers jours les propos du secrétaire d'État, Hervé Berville ont fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part de l'association Bloom devant la couver dans la cour de tout cela m'amène à quatre questions qui méritent des réponses claires pour lever les doutes qui demeurent sur nos pêcheurs hein si le Conseil d'État pointe inefficacité des dispositifs l'éloignement des dauphins sur les bateaux comme la situation acoustique par exemple. Le gouvernement envisage-t-il d'autres solutions de. Pouvez-vous nous dire précisément quelles sont les zones potentiellement concernés par l'interdiction de la pêche dans le Golfe de Gascogne. Détail important qui échappe au Conseil d'État trois si la pêche était effectivement fermé pour une durée cumulée de quatre mois, quelles indemnités pour sont prévues pour les pêcheurs. Quant à la et quand interviendront-t-elle et enfin pour vous et vous de clarifier les propos et les intentions de Monsieur le Ministre. À propos du plan d'action européen merci. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la la sénatrice. Alors vous parlez du du plan d'urgence c'est assez et comme vous le soulignez face au nombre important d'échouages de cétacés sur les plages de l'Atlantique à la suite de captures accidentelles dans les filets de pêche. Le gouvernement a mis en place un plan d'urgence en septembre dernier. Ce plan prévoit d'une part des équipements obligatoires comme des dispositifs de localisation d'effarouchement, et des caméras vidéo. D'autre part l'installation de ces dispositifs sur les 213 navires les plus actifs dans le Golfe de Gascogne. Dont 100 en caméra. C'est la première fois qu'un plan de ce type et mis en place aussi rapidement. Avec plus de 17 millions d'euros de financements publics un engagement des professionnels à agir ce plan et travailler avec les scientifiques, les ONG, les pêcheurs et doit tester des dispositifs qui permettront de concilier la pêche avec la présence de assez une évaluation de ce plan est prévue d'ici la fin de l'année 2024. Vous le soulignez aussi le Conseil d'État a rendu un jugement dans lequel il demande à l'État de garantir l'efficacité des mesures dès l'hiver prochain. Le gouvernement prend acte de cette décision. Ce jugement nécessaire nécessite pardon de réinterroger l'équilibre du plan d'urgence. Il va donc falloir remettre à plat ce plan d'urgence vous poser 4 questions. Je pense qu'il est encore trop tôt pour dire quelles mesures seront prises mais elles le seront les réponses seront étudiées dans tous les cas et concertée avec tous les acteurs je sais que mon collègue Hervé Berville associera les élus concernés afin de préserver bien sûr l'équilibre de ce plan et de ne pas opposer l'activité de pêche et la protection de l'environnement marin. Merci. Oh non non madame. Vous savez largement dépassé, merci. La parole est à Michèle bête. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues, j'ai souhaité interpeller le le gouvernement sur la question des chaudières au gaz. Nous sommes tous bien entendu interpellée par la nécessité de la transition écologique et énergétique, y compris les personnes en situation de handicap, y compris les jeunes notamment les jeunes du lycée Laënnec de Pont-l Abbé dans le Finistère qui nous écoute à l'heure actuelle. Mais il s'agit de faire attention à la manière dont tout cela va être réalisée il y a déjà eu, pour ce qui concerne les chaudières au fioul. Une interdiction d'installer. Ces chaudières dans les habitations nouvelles depuis. Juillet 2022 et il semblerait que la même interdiction se profile pour ce qui concerne la chaudière à gaz et ceci. Peut nous préoccuper parce que pour autant nous faisons aujourd'hui appel à du gaz d'origine fossile. Nous pensons en particulier en Bretagne que nous sommes en capacité de produire du gaz renouvelable du gaz vers Monsieur le Président. Et donc nous pensons que cela peut également d'ailleurs. Renforcer l'activité agricole et le permettre aux agriculteurs de d'obtenir de revenus complémentaires. Et c'est pourquoi j'ai souhaité savoir quelles étaient les intentions du gouvernement sur ce sujet des chaudières à gaz. Si Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le le sénateur, je vous prie d'excuser Agnès Pannier-Runacher. Qui est retenu en conseil des ministres. Comme vous le savez, le président de la République a fixé des objectifs très ambitieux en matière de transition énergétique. Être le 1er grand pays industriel à le se libérer de la dépendance aux énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Concernant le chauffage des logements. Depuis le début de l'année 2022, la réglementation environnementale R 2020 impose le recours à une part importante d'énergies décarbonnées pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les logements neufs. Cette première échéance s'est imposé aux maisons individuelles et s'étend progressivement au logement collectif en 2025 et dans les bâtiments tertiaires. Il n'y a donc à ce jour pas d'interdiction d'installation de chaudières à gaz dans les logements existants certaines aides tire. Les conséquences de cette évolution comme m'a pris une MaPrimeRénov pardon aide qui a permis de rénover près de 700.000 logements en 2022 mais qui ne subventionne plus l'achat de chaudières à fioul ou à gaz des solutions compétitives existe néanmoins réseaux de chaleur ENR système solaire. Et caetera. Enfin, s'agissant du biogaz. Je rappelle les ordres de grandeur en jeu aujourd'hui, nous avons consommé. En 2021, 480 TWh de gaz et nous avons actuellement une capacité d'injection dans les réseaux de 10 TWh de biogaz avec un gisement globale de biomasse qui restera limitée est fortement sollicité par ailleurs, vous le savez par l'industrie de la biochimie par exemple ou pour décarboner les secteurs qui n'ont que peu d'alternatives, comme l'aviation et le maritime. Donc réduire notre consommation globale de gaz n'est pas incompatible avec le développement fort du biogaz au service des secteurs et pour le cas où les alternatives au gaz sont elles limitées. Merci monsieur bête. Merci, madame la Ministre, de ces précisions mais. Je dois dire qu'il faut faire attention, d'une part parce que on a encore besoin du gaz beaucoup de d'habitation notamment dans le milieu rural sont chauffés au gaz, donc. Changer de mode de chauffage nécessiterait des investissements importants et tout le monde n'a pas les moyens d'une part et puis d'autre part la situation récente nous amène à à être prudents, c'est-à-dire de tout miser sur l'électricité risque de nous rendre particulièrement vulnérables et donc il est souhaitable de multiplier les sources d'approvisionnement énergétique sur le on ne veut pas se retrouver dans la difficulté, c'est le sens de mon intervention. Merci, cher collègue, la parole à Bruno Belin. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. La France est belle, riche d'un Patrimoine exceptionnel qui fait rayonner. Nos villes et qui. Aussi habille de façon le plus souvent magistral nos campagnes. Et bien souvent d'ailleurs en milieu rural, ce Patrimoine classés. Inscrits protéger non inscrits ou non classés appartient. Aux communes qui ont fait depuis des années des efforts. Vous avez vu le développement des petites cités de caractère des sites patrimoniaux remarquables et face à ça, les communes aujourd'hui ont bien du mal à entretenir ce Patrimoine historique exceptionnel bien du mal parce que les finances sont exemptes de vous le savez. Vous avez vous aussi exercer cette merveilleuse fonction de maire, vous le savez, parallèlement à ça pour monter les projets il y a la complexité d'un d'un dialogue. Parfois difficile. Il faut dire les choses avec les architectes des Bâtiments de France, on a besoin de parce qu'ils sont conseil parce qu'ils sont sachant parce que ils vont apporter évidemment aux élus. Une orientation souvent importantes, mais le risque de surcharger les prescriptions, les exigences parfois les le manque de cohérence parce que. Évidemment comme tout fonctionnaire il y a une rotation des postes. Font qu'aujourd'hui, les communes, les maires ne comprennent pas ce qui leur arrive et ne peuvent pas assumer de travaux importants sur des projets. Essentiels pour leur commune est essentielle pour l'économie locale parce que ça fait travailler les entreprises du secteur. Alors Madame la Ministre. Je voudrais savoir comment il serait possible. Voilà d'imaginer. Évidemment une concertation en tout cas un dialogue une écoute pour que mère et ABF s'entendent pour que les projets des communes puisse se faire. Merci, cher collègue, la parole est Madonna Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le le sénateur. Vous poser un problème important, c'est la conservation de notre Patrimoine la mise en valeur de notre Patrimoine dans toutes les communes de France des plus grandes aux plus petites

Et qui apporte des conseils qui sont des conseils parfois de de enfin que souvent de très très bonne qualité, bien sûr. Ces espaces remarquables que nous devons protéger c'est environ 6% du territoire national et ça contribue vraiment au rayonnement culturel à l'attractivité touristique et économique de la France la protection de ces espaces a donc été confiée par le législateur. Aux ABF qu'il exerce grâce à ce qu'on appelle l'avis conforme. Alors vous l'avez souligné, protéger et préserver notre Patrimoine doit se faire en bonne Intelligence avec les élus locaux et je veux rappeler que la vie de la BF et toujours rendu au cas par cas en fonction de chaque projet et des enjeux locaux et contrairement à ce qu'on pourrait croire cette collaboration fonctionne quand même bien puisque, sur plus de 500.000 dossiers de travaux instruit chaque année par les ABF. Seuls 7% en moyenne, font l'objet de l'avis défavorable. Lorsque un premier projet refusé il est souvent suivi d'un projet modifié et in fine et qui est accepté les ABF exerce en effet plus de 200.000 Conseil chaque année pour permettre de favoriser des solutions plus adaptées à la conservation du du Patrimoine et la mise en valeur du Cadre de vie et en cas de désaccord. Une procédure d'appel existe le porteur de projet et l'autorité compétente. Pour délivrer l'autorisation peuvent contester un refus d'autorisation et de prescriptions de la bf devant le préfet de région et ils peuvent ensuite saisir les juridictions administratives. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup ça, ça fait toujours perdent du temps dans les dans les dans les dossiers dont vous le voyez, je crois qu'il faut les prendre pour des partenaires et des partenaires fiables.

ils sont sous l'autorité des préfets de région, je crois qu'il faudrait les placer sous l'autorité des préfets de département, parce qu'on a un corps préfectoral exceptionnelle en France, qui connaît bien, il y a un an le sujet local et puis effectivement à la fin, il faudrait que le dernier mot reviennent au maire. Merci madame maladie. Merci monsieur Laurent Bureau. Merci monsieur le président, madame la ministre, ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux. Afin d'éviter un trop long procès pénal des mesures alternatives peut être prise par le procureur de la République. L'objectif étant d'assurer rapidement la réparation du dommage causé de mettre fin bien sûr à l'infraction mais aussi de sensibiliser l'auteur des faits aux conséquences de ses actes. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2021, améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, le procureur de la République peut également demander à l'auteur des faits de verser une contribution dite citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes avec laquelle le tribunal a signé une convention. Le montant de cette contribution dans le monde un maximum est de 3000 euros est alors fixée par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur. Cependant, la principale victime et parfois l'environnement. Le département du Gard est un particulièrement concerné par le réchauffement climatique sécheresses, feux mais aussi inondations. Je regrette que les associations agréées de défense environnementale ne puisse être bénéficiaire de ces contributions citoyennes. Vous l'aurez compris, il me semblerait pertinent qu'à l'occasion d'une incivilité, entraînant une pollution une infraction aux règles de l'urbanisme ou encore en comportements à risque en matière d'incendie. Ces associations puissent donner davantage de sens à la sanction pénale, madame la Ministre, seriez-vous d'accord pour qu'elle puisse recevoir ces contributions citoyennes et si oui comment leur permettre je vous remercie. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le. Le sénateur vous poser une question importante sur ce problème majeur de l'indemnisation du dommage causé en matière environnementale. Alors dans les suites de la jurisprudence Erika la loi du 8 août 2016 a consacré la réparation du préjudice écologique, encadré par les articles 12 46 et suivants du Code civil, bien que de nature civile la notion de préjudice écologique a légitimement vocation à être convoqués au stade du procès pénal par les parties civiles, dont les associations agréées de protection de l'environnement qui entendent obtenir une indemnisation. Ce qui correspond à l'analyse qu'en fait la Cour de cassation. Outre les associations de défense de l'environnement bénéficient de la convention judiciaire d'intérêt public environnementale la CEJ Créé par la loi du 24 décembre 2020 qui leur permet d'obtenir réparation du préjudice écologique, là où la procédure de transaction pénale environnemental autorisées seulement le paiement d'une amende transactionnelle ce ce cette CJ IPE permet une indemnisation accéléré sans attendre la condamnation définitive de l'entreprise par un tribunal ou une cour d'appel pouvant prendre plusieurs années. La victime pourra être informé par le parquet avant la convention afin de pouvoir transmettre tout élément de nature à établir son préjudice et la réparation doit intervenir dans un délai maximal de nom à compter de la signature de la CIJ C'est un réel succès 9 conventions ayant été conclu devant depuis sa création, certaines ayant donné lieu au versement de dommages et intérêts significatifs à des associations, donc le dispositif législatif actuel offre donc toutes les possibilités effectives pour les associations de défense de l'environnement, d'obtenir réparation tente devant le tribunal correctionnel que dans le cadre de ces fameuses C.

Ma question puisque c'était de la part des parquetiers gardera de Nîmes et d'Alès qui disent que dans le cadre des ça alternative à la poursuite, c'est-à-dire que l'eau d'aller au procès pénal il pourrait prononcer. Cette amende. Citoyenne d'un maximum de 3000 euros. Voilà, là vous me parlez. Dans le cas d'un procès pénal ou les associations environnementales peuvent être indemnisés je tout à fait d'accord avec vous, c'est une alternative se reposer. Au procès pénal. Et ça serait bien que pour des petites infractions en matière d'environnement, cela puisse être le cas. Merci madame Sylviane Noël. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre à travers la création du service d'accès aux soins, le sas 74 il y a maintenant 2 ans. La collaboration entre tous les acteurs médicaux de Haute-Savoie a permis d'améliorer la régulation des appels d'urgence grâce à l'action de plus de 350 médecins généralistes. Le 15 et les services d'urgences constate déjà une nette amélioration en termes d'afflux de patients. Actuellement, le financement national prévu par le sas permet de valoriser la participation des médecins ce dispositif et valorise ainsi les efforts faits pour recevoir des patients n'ont connu des cabinets. Or, la directrice de la CPAM de la Haute-Savoie a unilatéralement décidé en février dernier qu'elle refuserait de financer désormais l'application de la majoration pour SNP de 15 euros par consultation si le patient n'a pas été au préalable, dirigée par le Centre 15, cette décision injustifiée et incompréhensible, va à l'encontre de l'instruction ministérielle de juillet 2022 et aboutira à engorger inutilement le centre 15. Alors que le département de la Haute-Savoie subit déjà une double peine à travers d'une part les nombreuses déserts médicaux dans ces zones rurales et de montagne et d'autre part la fuite incessante des professionnels de santé en Suisse voisine, où les salaires sont bien plus élevés. Cette décision technocratique et irresponsable et réduit à néant les progrès obtenus sur le terrain depuis plusieurs mois par ces professionnels. J'en appelle donc à l'arbitrage du gouvernement pour s'opposer à cette nouvelle décision de la CPAM de Haute-Savoie qui constitue, avec la révision du barème kilométrique des infirmiers libéraux, un coup dur insupportable pour notre système de soins déjà en grande souffrance. Je vous remercie. Merci monsieur le le président, madame la la sénatrice. Votre question porte donc sur la situation du service d'accès aux soins de Haute-Savoie. Pour lequel la la CPAM ne verse pas au au médecin de majoration de 15 euros

pour les équipements, le Fonds pour la modernisation de l'investissement en santé et pour la valorisation de la participation des médecins l'enveloppe des soins de ville. Alors j'ai pas tout à fait la même lecture que vous de l'instruction du 10 juillet 2022. Puisqu'elle a instauré une majoration de 15 euros pour tout acte effectué par un médecin à la demande de la régulation du SAMU ou du sas pour un patient hors de sa patiente médecin traitant dans la limite de 20 consultations hebdomadaires. Par conséquent, la position de la CPAM 74 de ne pas verser cette majoration. Systématiquement et pour, et notamment pour les consultations qui n'ont pas été régulé par le sas SAMU et justifiée. Elle ne relève en rien d'une décision arbitraire ou unilatérale c'est une position qui est partagée par l'ARS Auvergne Rhône-Alpes. Aujourd'hui l'enjeu principal est de permettre à la montée en charge de l'activité du sas pour l'amélioration pour améliorer l'accès aux consultations Nous avons conscience que cela devra passer par une plus grande adhésion des médecins effecteur à la plateforme, seules 146 d'entre eux étaient inscrits début avril l'ARS et la CPAM 74 partagent la même vision sur cette nécessaire évolution et Monsieur le Ministre de la Santé et de la prévention l'avait annoncé dans ses voeux, une mission d'accompagnement au déploiement des sas va très prochainement être mis en place donc évaluation monter en puissance accompagnement. Merci, madame la Ministre, pour votre réponse. Qui ne satisfait pas vraiment vous vous en doutez. De grâce, faites confiance aux acteurs de terrain qui mène des expérimentations intéressantes et qui font preuve de leur efficacité.

La parole est à madame Darcos. Ma question s'adresser au ministre de la santé, la prévention, madame la Ministre. Le Centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes est réputée pour l'excellence de son offre de soins. Ce n'est pas un hasard si le président de la République a choisi cet établissement pour y présenter ses voeux aux acteurs de la santé le 6 janvier dernier. Fortement soutenu par les collectivités territoriales, département de l'Essonne agglomération Grand Paris issus des villes d'Evry-Courcouronnes il poursuit une triple mission de soins d'enseignement et de recherche. Pivot du groupement hospitalier de territoire Île-de-France sud avec le Centre hospitalier Sud Essonne Dourdan Etampes et le centre hospitalier d'Arpajon il assure une médecine de proximité et de recours dans une quarantaine de spécialité ainsi qu'une importante activité d'urgences adultes gynécologique et pédiatrique. L'établissement est actuellement doté de de services hospitalo-universitaire en de diabétologie endocrinologie. Et en neurologie, en lien avec l'INSERM, les facultés de médecine et de pharmacie Paris-Saclay et le Génopôle, 1er biocluster français, il met en place depuis 2018 des actions destinées à renforcer la continuité recherche fondamentale soin et à faciliter l'interface investigateurs patients. Il veille aussi à favoriser l'innovation hospitalière et l'intégration des médecins et pharmaciens dans les équipes de recherche du site et à créer un écosystème favorable aux carrières hospitalo-universitaire. Au regard de l'excellence KT caractérisant l'activité les personnels du Centre hospitalier Sud francilien. Il serait parfaitement légitime de lui accorder les moyens de poursuite de poursuivre son Entendez-vous accéder à cette demande qui permettra de maintenir une offre de soins de pointe accessible et public tout en développant les activités de recours et d'excellence sur le territoire de l'Essonne. Je vous remercie. Merci monsieur le président, madame la la sénatrice. Sur le le ministre François Braun m'a m'a chargé de vous répondre et de vous dire que bien sûr la place et ce qu'elle était la place essentielle et l'excellence du Centre hospitalier Sud francilien. En Île-de-France. Alors vous l'avez dit de spécialités de l'hôpital sont aujourd'hui. Des spécialités universitaires landau créneau diabétologie et la neurologie avec 5 post-universitaire rattaché à la faculté de médecine de l'université Saclay. Ainsi le CHSF est un hôpital qui dispose donc de praticiens universitaire, avec des tentes dédié aux activités d'enseignement et de recherche en complément de leur activité clinique c'est post-universitaires favorise l'attractivité de ce centre hospitalier et il contribue au rayonnement de la recherche et de l'innovation sur le territoire en lien avec le Genopole université d'Evry Paris Saclay les écoles d'ingénieurs du territoire IRBA l'INSERM donc tout un écosystème. Particulièrement intéressante dans l'activité de recherche avec des axes stratégiques du projet médical du CHSF. La croissance dynamique de la recherche clinique. A permis en 2021 de mener, près de 210 études et d'inclure 907 patients. Donc à partir de ce constat et bien bien sûr l'ARS ce soutien avec le doyen de la faculté de médecine les initiatives de développement de cet univers si tu. Starisation. Mon pas facile à dire et dans les jours à venir, elle organisera à ce titre une réunion avec les élus, le doyen de la faculté de médecine, la direction, la présidente de la communauté médicale du CH SF pour avancer sur une nouvelle étape. D'univers site Ariza Sion cela pourrait notamment passer par l'attribution de nouveaux postes universitaires dans les disciplines déjà concernés. Et et et le cas échéant, le développement de nouvelles disciplines universitaires en tout cas l'action de l'ARS portera vraiment. Sur l'attractivité de l'hôpital aussi pour les internes qui sont souvent la base de tout développement de recherche dans en clinique. Si Madame Darcos ce quelques secondes. Non mais écoutez remercier le gouvernement en effet le 6 janvier dernier on avait pu. Exprimer cette demande au président de la République et et à la présidence, la directrice de l'ARS en en Direct et donc en effet je je sais qu'il y a cette réunion très prochainement et donc j'espère qu'elle sera suivie d'effet. Merci la même ici. La parole est à monsieur Théophile. Madame la ministre, ma question s'adresse au ministre de la Santé de la prévention. Le 5 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles. Ces années de procédure n'auront pas suffi à établir clairement les faits et a condamné les responsables de ce scandale sanitaire. Il reste au-delà des procédures de justice que cet insecticide a contaminé les sols les ou les cultures les productions animales et plus grave encore les corps, selon Santé publique France, plus de 90% de la population adulte de Guadeloupe et de Martinique est contaminée. Les conséquences sont terribles. Le lien entre le cancer de la prostate est une ex-une sous-Exposition au chlordécone a été récemment établi les Antilles détiennent, vous le savez, un triste record mondial avec une incidence. Plus de 2 fois supérieur à la moyenne de l'Hexagone. Les femmes elles-aussi pourrait ne pas être épargnée si le lien entre le cancer du sein et cette molécule, n'a pas été formellement établi. Il n'en demeure pas moins que la précocité de de l'incidence interroge en Guadeloupe, près de 20% des cancers du sein sont ainsi diagnostiqué chez les femmes âgées de moins de 50 ans face à ce constat de pistes se dégagent. Chez les hommes de plus de 45 ans un dépistage organisé, à l'instar du programme national de dépistage du cancer colorectal aurait pour effet d'augmenter la démarche de prévention, de prévention et permettrait de mieux recourir à d'autres examens chez les femmes, il conviendrait d'abaisser l'âge cible du dépistage organisé du cancer du sein pour offrir aux guadeloupéenne et martiniquaise les mêmes chances que dans l'Hexagone. Je serai heureux Madame la Ministre, de connaître la position du gouvernement sur ces différentes propositions. Le plan chlordécone quatre est un plan ambitieux auquel je m'associe pleinement. Il nous faut cependant aller beaucoup plus loin, je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le sénateur. Oui le les conséquences sanitaires de l'utilisation du chlordécone sont un sujet de préoccupation constant pour le le ministre, le ministre et c'est pourquoi compte tenu de la sur-incidence. Du cancer de la prostate en Guadeloupe et Martinique. Il a été mis en place des actions renforcée de sensibilisation des des populations et des professionnels. Le Centre régional de coordination de dépistage des cancers de la Guadeloupe anime des séances d'information et de sensibilisation au dépistage dans les communes au sein des quartiers les plus défavorisés éloigné où la présence des soignants est plus faible dans une logique de proximité. Ces séances organisées en liaison étroite avec les maires, les professionnels de santé du territoire rassemble de plus en plus de personnes et c'est, c'est important de le dire aussi, le cancer de la prostate est reconnu depuis 2021 comme l'une des maladies professionnelles pouvant être liés à une exploration une Exposition aux pesticides dont la chlordécone, les premières indemnisations des des victimes commencent à être versées aux Antilles et de nombreuses mesures sont engagés pour réduire l'Exposition de la population mais nous devons continuer et continuer à faire mieux et notamment dans les rendez-vous de prévention qui vont être mis en place pour la population générale, mais qui seront un vrai moment important pour pouvoir porter ses actions de prévention dans les Antilles sur ce sujet de la chlordécone ses rendez-vous de prévention des âges 40 45 ans et 60 65 ans ils vont vraiment permettre d'aborder avec les patients dans ces territoires concernés. Le dépistage des cancers. Ceux de la prostate et ceux du sein et lors des premiers comités de suivi de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. 2021 2030. En décembre dernier, l'importance de la prévention des dépistages a été rappelé, et nous allons renforcer toujours la recherche dans le domaine des dépistages pour requestionner les bornes d'âge des dépistages organisés et proposer des recommandations pour les personnes qui n'en relèverait pas. Merci la parole est à Philippe mouiller. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Créé par la loi du 11 février 2005. La prestation de compensation du handicap, vise à permettre aux personnes en situation de handicap de financer des aides de différentes natures dans le but d'assurer leur autonomie. L'article 3 de la loi du 6 mars 2020, visant à améliorer la PCH dont j'ai été l'auteur donc je la connais bien introduit dans le code de l'ex-sociale et des familles a pour objectif d'améliorer les contrôles d'effectivité de la PCH. Ces contrôles représente une étape importante dans le parcours d'accès aux droits des personnes en situation de handicap et sont très souvent source d'inquiétude et de difficulté pour celle-ci. Or il s'avère que les dispositions relatives aux contrôles sont appliquées de manière différente selon les territoires. Alors que l'article L 245 5 du code de l'ex-sociale et des familles prévoit que la période de référence ne peut être inférieure à six mois, les bénéficiaires de la PCH constate que sur certains territoires. Les contrôles se font sur des périodes inférieures ou qu'ils ont été ramenés à six mois sur des territoires sur lesquels il s'effectuer sur des périodes allant jusqu'en un an. L'esprit de la loi du 6 mars 2020 n'est donc pas respecté ou minorée. En effet, la souplesse de la période de contrôle introduits par ce texte avait pour objectif une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et donc, je pense notamment qu'il y a souvent des écarts entre un plan d'aide et sa mise en oeuvre effective, notamment pour des raisons de vacances pour des raisons de maladie pour des phases de répit. Cette problématique est forcément moins importante qu'on le contrôle s'effectue sur une période plus longue au minimum de six mois. Au delà de la la cette PCH cette ça se passe de contrôle finalement est source d'importantes incompréhension et les personnes en situation de handicap, hé bien ne comprennent pas pourquoi la loi n'est pas respectée. Je voudrais Madame le Ministre connaître votre point de vue et surtout que vous entendez faire pour améliorer cette effectivité ces contrôles. Merci, madame la Ministre. à la prestation de compensation du handicap. Alors je veux rappeler que la PCH, vous le savez bien sûr est une prestation en nature. Qui vise à couvrir les frais que supportent une personne en raison de son handicap et qui est essentiel pour leur autonomie et que, à sa création la PCH a répondu à une forte demande des associations en mettant en place une prestation très personnalisé. Alors ces contrôles d'effectivité confiée confiée aux conseils départementaux permettent de garantir que ces aides serve réellement la personne dans la compensation de son handicap. Toutefois ces contrôles ne s'applique pas dans certaines situations,

L'introduction de cette période de contrôle par la loi du 6 mars 2020, visant à améliorer l'accès à la PCH. Sur une durée suffisamment longue apporte plus de souplesse pour les personnes. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a communiqué à plusieurs reprises au MDPH et surtout aux conseils départementaux sur la durée minimum de six mois pour le contrôle d'effectivité. La CNSA a aussi rappelé que le report d'heures d'un mois sur l'autre est possible sur cette période de 6 mois pour des heures effectuées en PCH aide humaine. Ainsi la fonction en fonction de leurs besoins ou de leurs souhaits, les bénéficiaires peuvent faire fluctuer librement. Le nombre d'heures d'aide humaine et qu'elle mobilise la CNSA se fera à nouveau le relais de cette disposition importante pour les personnes en situation de handicap via la documentation qu'elle élabore et la diffus et diffuse dans le cadre de ses missions de pilotage et d'animation. Je dois dire que depuis 2020 nous avons permis une réelle harmonisation des pratiques pour les bénéficiaires de la PCH dans tous nos départements et que l'harmonisation et équité sont pour moi des principes fondateurs de la prise en charge des personnes en situation de handicap et que nous continuerons à y travailler. Merci monsieur quelques secondes non. La parole est à madame. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre dans mon département, la Haute-Vienne il ne se passe pas une semaine sans que la presse locale se fasse l'écho de classe sans enseignant, dans le 1er degré. Lorsque j'ai interrogé le ministre de l'Éducation nationale sur la carte scolaire en janvier dernier, près d'une centaine de classe n'avait pas d'enseignants. Ce nombre élevé était dû en grande partie à l'épidémie de grippe. Mais bien que celle-ci soit terminé. Le nombre de classes sans enseignants restent encore particulièrement élevé une quarantaine il y a 15 jours et plus d'une trentaine encore la semaine dernière. La situation est telle que dans certaines écoles et classes n'ont pas cours en début ou en fin de semaine, d'autres n'ont pas d'enseignants depuis même plus d'une semaine. Quant aux enfants sans mettre, ils sont au mieux répartis dans les autres classes qui compte dès lors bien souvent 30 voire 35 élèves et lorsque ce n'est pas possible une garderie est alors improvisé. Voilà le quotidien de nombreux enfants. Enseignants, parents d'élèves et élus de la Haute-Vienne. Ceci s'explique par l'insuffisance du nombre de remplaçants disponibles, les 138 enseignants de la brigade de remplacement sont en effet déjà tout son poste devant les élèves. Il n'est pas acceptable que la la scolarité des enfants soient ainsi perturbée par la faiblesse des moyens humains et financiers accordés à l'éducation nationale. Ma question est donc simple, quelles mesures entendez-vous prendre pour garantir la qualité et la continuité du service public de l'éducation nationale dans les écoles de la Haute-Vienne. Je vous remercie. Si Madame la Ministre. Merci monsieur le le président, madame la la sénatrice le remplacement des professeurs absents constitue une une priorité du service public de l'éducation nationale, alors nous devons répondre à des objectifs de continuité pédagogique. De garantie de la qualité du service rendu aux élèves et aux familles dans les écoles, collèges et lycées. À la rentrée 2022 près de 30.000 personnels en équivalents temps plein sont mobilisés pour le remplacement dans le 1er degré, soit 9% des effectifs enseignants. Outre des mesures sont prises pour déplacer lorsque cela est possible les formations et autres obligations des enseignants hors du temps devant les élèves, par exemple le mercredi après-midi. De plus, un logiciel d'aide au remplacement est en cours de déploiement national dans les académies pour réduire le temps de traitement donc de latence entre l'expression du besoin et le remplacement effectif en ce qui concerne l'académie de Limoges, la baisse démographique constaté depuis plusieurs années, moins 5000 élèves de 2018 à 2023, dont moins de 1500 dans dans la Haute-Vienne. Allié à la non-suppressions de postes a permis une hausse régulière des taux d'encadrement des élèves du 1er degré sur l'académie. Cette progression se poursuivra à la rentrée 2023, il n'en demeure pas moins que la situation locale que vous évoquez reste difficile. Depuis le mois de mars, le département de la Haute-Vienne connaît des difficultés pour couvrir les remplacements long. Avec dans certains cas des remplacements opérés de enfin de manière discontinue par des enseignants différents et effectivement depuis le 31 mars. On peut évaluer à une trentaine de classe non remplacés par jour donc. Soyez certaine que l'Académie restent très mobilisés pour répondre aux besoins et travaille à la fidélisation des viviers d'enseignants contractuels et à la détection de nouveaux viviers. Pour accompagner ces remplacements qui sont bien sûr une préoccupation majeure de l'Académie, mais aussi du ministre de l'Éducation nationale. je vous remercie. Madame la Ministre ne de prendre particulièrement à coeur cette préoccupation parce que. On nous dit évidemment qu'il y a les moyens mais le souci c'est que sur le terrain, personne ne voit les choses de cette façon les absences d'exceptionnel. Elles deviennent la norme et ça c'est pas possible et c'est pas la, la carte scolaire qui est prévu pour un, pour la rentrée qui va qui va arranger les choses. Se pose aussi la question n'a pas été vous mais de l'attractivité du métier puisque selon le l'inspection académique, il y aurait 12 recrutement possible aujourd'hui et il y a pas de candidat. Donc nous avons là un vrai souci. RC Monsieur Gillet. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre les missions locales présidée par les représentants des collectivités territoriales organise le service public de l'accompagnement et de l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans sans distinction. Elle pilote l'élaboration et la mise en Oeuvres d'un projet territorial et partenariale favorisant l'accès des jeunes à l'autonomie en partant de leurs ressources. C'est donc naturellement qu'elles se sont rendus aux concertations sur le plein emploi organisé par Emmanuel Macron alors candidat à son second mandat. Les missions locales sont depuis en attente d'un retour. Le rapport du Haut commissaire pour l'emploi doit être rendue dans les prochaines semaines. Mais les inquiétudes se font grandissantes en effet si elle partage l'idée d'une coopération renouvelée entre les différents acteurs. Elles craignent une mise en concurrence entre leurs entités et celle de France travail anciennement Pôle emploi. Il serait donc dommageable qu'elle change d'appellation pour être ramenée à un pôle emploi jeune avec une mise sous tutelle. En effet, les missions locales ne saurait être réduite à leur seule mission d'insertion professionnelle. Elle touche également problématique de logement de l'accès aux soins handicap Loisirs Mobilité finalement tous les remparts à l'exclusion sociale. C'est ce qui fait leur originalité reconnue sur le plan européen. Ainsi l'algorithme d'orientation comme point d'entrée obligée pour le 1er contact dans l'accueil des jeunes pose un grand nombre de questions puisqu'il risque d'entraîner une stigmatisation supplémentaire. La mixité est un atout qui permet à toutes et à tous de vivre ensemble et d'avoir pour horizon politique, l'égalité des chances. Seule l'entretien conseil permet de discerner les profils et les problématiques Madame la Ministre l'intégration des missions locales dans France travail provoquera une perte d'identité et un affaiblissement de la singularité de ce réseau. Comment les rassurer. Quelles garanties pouvez-vous leur donner. Madame la ministre. Merci monsieur le le président monsieur le le sénateur vous dites votre attachement aux missions locales, sachez que le gouvernement est aussi très attaché aux missions locales Vous avez rappelé l'implication et l'utilité des missions locales pour aller vers les jeunes les plus éloignés de l'emploi et les accompagner dans leur insertion professionnelle. Alors nous partageons votre constat et nous nous réjouissons du travail d'accompagnement de qualité réalisé par les missions locales et de fait elles continueront à jouer ce rôle et pourront devenir France travail jeune. D'ailleurs, ça aura plus de signification en terme. Auprès des jeunes que Mission locale qui quelquefois. Sémantiquement. Peut paraître un petit peu éloigné. Moi je crois que l'État a témoigné de sa confiance aux missions locales avec le déploiement du contrat d'engagement jeune, l'appel à projets pour les jeunes, dits en rupture mais aussi l'accompagnement de jeunes en situation de handicap et et je sais dans la mission que j'ai de de quoi je parle. Mais France travail je ne contribuera aux côtés de France travaille à élaborer la feuille de route annuelle pour le public jeune sur chaque territoire cette feuille de route ou co-, construite avec les acteurs concernés proposera un retour sur les résultats, année après année un diagnostic de la situation actuelle et détaillera les objectifs communs en matière, en matière de repérage d'accompagnement et de retour à l'emploi des jeunes. Elle permettra enfin d'animer l'écosystème de l'insertion locale en décrivant des partenariats à mobiliser et les moyens à y associer les comités France travail locaux co-coprésidé par l'État et les collectivités territoriales examineront ensuite ces feuilles de route ce schéma de gouvernance collectif intégrera sans modifier la contractualisation entre les missions locales et ses financeurs le conventionnement directe avec l'État et les collectivités. Donc France travail jeune pourra prendre l'initiative pilotée et être garant des projets directement auprès de l'État et des collectivités dans le cadre de contractualisation et de feuille de route commune donc. Si. Merci, madame la Ministre quelques secondes monsieur Gillet. Madame la Ministre quand on change de nom perd souvent de cultures et d'identités. Mais moi je vous propose, qui tient un protocole qui soit mis en place, de discussions et de négociations pour cette éventuelle intégration dans la dimension France travail ça permettrait de rassurer l'ensemble des acteurs. Je vous en remercie. La parole maintenant Monsieur Jean-Jacques Panunzi. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Madame la Ministre, la Corse qui est l'île la plus boisée de Méditerranée. Connaît chaque année des incendies importants et ravageur et plus seulement durant les 2 mois de l'été. Le réchauffement climatique est devenu une évidence et ses conséquences sur l'inflammabilité de la végétation méditerranéenne se traduisent par des feux au démarrage foudroyant et au développement tellement rapide que la présence de moyens aériens sur place tant en alerte au sol qu'en alerte au vol est devenu incontournable. Le Canadair 415 et l'outil adéquate pour intervenir en cadence élevée sur les départs de feu avant qu'il ne se propage fortement. Et remplit ses soutes d'un total de 6000 litres d'eau et de retardant 12 secondes et transporte sa charge à la vitesse de quatre kilomètres à la minute. À ce jour, la sécurité civile possède une flotte vieillissante d'11 appareils tous regroupés à Nîmes donc un peu plus éloigné de la Corse que lorsqu'il était basé à Marseille avec 1h30 de trajet pour gagner l'Lille. Pendant la saison estivale, ils sont repartis entre les Landes, la Provence et la Corse cette dispersion est régulièrement remplacées par des regroupements lorsque des incendies sévère incontrôlable conduisant à l'abandon temporaire par les appareils de leur secteur d'affectation. Des gains substantiels peuvent être réalisées dans le cas d'une gestion globale des moyens avec moins d'heures de vol et de trajet, une capacité d'intervention plus rapide et une bonne prévention. L'efficacité des intervenants au sol. La dégradation climatique justifie de régionaliser les moyens de lutte contre les incendies et d'instaurer une permanence des moyens via des unités de bombardiers d'eau basés en Corse pour pouvoir disposer d'une protection optimale face aux incendies. Ces unités se substituerait à celle affrété depuis le continent et aux de tracteurs basée à Bastia. Madame la Ministre, dans le contexte actuel d'urgence climatique. Souscrivez-vous à cette proposition d'instaurer une présence permanente d'unités de bombardiers d'eau en Corse afin de prévenir les feux et d'intervenir dans les meilleurs délais. Dès qu'un incendie est identifié. c'est à vous. Bonjour monsieur le président et. Merci monsieur le sénateur Panunzi. Le ministère de. L'Intérieur et des Outre-mer dispose d'une flotte actuellement composée de 12 canadairs canadairs bombardiers d'eau amphibie de 7 Dash 8 bombardier d'eau et de 3 Beach 200 1/8ème d'âge viendra compléter ce dispositif au 1er juin 2023, la flotte de Canadair sera renforcé par deux appareils financé par l'Union européenne et 2 appareils supplémentaires acquis sur fonds propres, le président de la République a par ailleurs décidé du remplacement de la flotte de Canadair par des appareils de nouvelle génération, de la sécurité civile de Nîmes-concentre les flottes avions et hélicoptères Les hangars dédié à la maintenance, les unités de formation ainsi que les services de soutien cette centralisation des moyens permet une meilleure rationalisation des coûts de fonctionnement des infrastructures ainsi que des moyens humains et une meilleure efficacité et adaptabilité de notre organisation, elle se concrétise durant la saison feu par le prépositionnement d'avion suivant les risques, il est à noter que la Corse dispose de manière spécifique et unique d'un site de détachements opérationnels activé durant toute la saison feu et armé et armé par 2 avions bombardiers d'eau. Enfin s'agissant des pilotes d'avion ce métier très fortement à risques nécessite un haut niveau d'entraînement tout au long de l'année pour maintenir un niveau socle d'entraînement et obtenir ainsi durant l'été, au degré de performance et de technicité. Les pilotes de la sécurité civile sont pour beaucoup issus de carrière militaire dans lesquels ils ont déjà acquis une grande expérience conscient cependant de la nécessité de fidéliser ses pilotes. Le ministre de l'Intérieur a signé mardi dernier, mardi 11 avril, un protocole d'accord avec les organisations syndicales pour valoriser ses métiers à risques et fidéliser ces personnels. C'est un accord sans précédent dans l'histoire de la sécurité civile, je vous remercie. Merci la parole est à madame Vermeillet. Merci monsieur le président, madame la ministre, depuis 2018, les policiers municipaux peuvent s'équiper de caméras individuelles afin de filmer certaines interventions. Le décret du 2 novembre 2002, pris en application de la loi numéro 2021 tirer 646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés vient renforcer cette disposition en précisant qu'il est désormais possible pour ces policiers de transmettre en temps réel à leur commandement, les enregistrements vidéo réalisés lors de leurs interventions. Il est également possible d'accéder directement aux images et de conserver ponctuellement un moyen permettant d'identifier les auteurs et de caractériser les faits ces évolutions contribuent grandement à faciliter l'émission elles ont également fait la preuve de leur efficacité pour limiter les agressions et insultes dont peuvent être victimes les policiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions en zone rurale majoritairement dépourvu de polices municipales ou intercommunales, la loi prévoit une expérimentation jusqu'en novembre 2024. Des caméras individuelles pour les gardes champêtre. Mais les agents de surveillance de la voie publique qui assurent des missions de surveillance du domaine public et sont exposées à ce titre aux mêmes actes d'incivilité que leurs collègues policiers ne peuvent être équipés de ces dispositifs aussi afin de permettre à l'ensemble des agents municipaux ayant ses missions de surveillance, de pouvoir réagir face aux actes malveillants dont ils peuvent être les victimes. Je vous demande Madame la Ministre dans quelle mesure une expérimentation de possession de caméras piétons au bénéfice des agents de surveillance de la voie publique pourrait être mise en oeuvre. Merci, merci madame la ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Vermeillet. Les agents de surveillance de la voie publique ou. ou. ASVP sont des agents communaux titulaire ou contractuel, chargé d'une mission de police. Vous proposez de leur permettre l'usage de caméras individuelles toutefois ces caméras porte atteinte au droit. Au respect de la vie privée des personnes filmées leur usage doit à ce titre être particulièrement encadré et strictement proportionnées aux finalités poursuivies et aux missions exercées. L'application du droit de la protection des données à caractère personnel conduit ainsi à en limiter l'attribution à des catégories de personnel et pour des situations strictement délimité. En effet si Lula l'usage des caméras individuelles, a été autorisée pour certaines catégories agents c'est en raison du caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée, eu égard aux buts poursuivis et aux fonctions exercées dans le cas présent une extension du dispositif des caméras mobiles au ASVP ne me paraît pas répondre à un besoin impérieux impérieux ni reposer sur des motifs pertinents et suffisants car contrairement aux policiers municipaux et aux garçons prête les ASVP dispose d'un Champ d'intervention particulièrement restreint. Exerçant principalement des missions relevant de la police de la circulation et ne dispose d'aucune prérogative de police judiciaire ainsi leurs compétences de verbalisation est très limitée, notamment au domaine du stationnement limité. À la propreté des voies et espaces publics et limitée à la lutte contre le bruit. Dans ces conditions, ces agents ne peuvent être regardées comme exerçant des missions de nature à justifier qu'il soit autorisé à filmer leurs interventions au moyen de caméras individuelles et même à titre expérimental je vous remercie. Merci, madame la Ministre, pour. Venir en aide aux mères et aux aux forces de sécurité. Par les temps qui courent, merci. Si la parole est à monsieur patients. Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues. La Guyane est devenue le département le plus criminogène et le plus violent de France. Les faits d'armes, agressions, crimes meurtres s'multiplient. Plus une seule partie du territoire n'est à l'abri de la violence et plus personne non plus. L'assassinat du gendarme Arnaud blanc en plein coeur de la forêt amazonienne qu'est la triste démonstration et je tiens ici à rendre hommage à ces hommes qui se dévouent jusqu'à donner leur vie pour la sécurité de leurs concitoyens. Madame la Ministre. L'État se doit d'assurer la sécurité de tous. Partout dans les grandes villes mais aussi dans les petites communes. Elles aussi confrontées à cette insécurité galopante. Lors de des Assises de la sécurité en Guyane, en septembre 2022, à Cayenne. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des renforts de gendarmerie sous forme de brigades nouvelles pas crier. Six mois après qu'en est-il. Quand ces nouvelles brigades seront. Et où il y a urgence. Je pense notamment à la brigade de Manas qui n'est plus suffisamment dimensionné pour couvrir son aire géographique d'intervention. Mais aussi j'ai avoué Charvin hawala y aller ma peau. Plus de 200 kilomètres de voies nationales et territoriales. Je pense aussi aux communes de Roura et de Montsinéry grandes. De plus en plus frappés par les crimes et délits et qui, elle aussi, vous en solliciter à juste titre. Alors Madame la Ministre quand se rend-elle installer ces nouvelles brigades. Si Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur patients depuis 2017, le président de la République fait de la sécurité du quotidien. La priorité de son mandat, cette ambition s'est traduite par la création dans votre département de 94 postes de gendarmes depuis 2017 au profit du commandement de la gendarmerie de la Guyane. Cet effort va se poursuivre. Dans le cadre d'une loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur pour améliorer la sécurité des Français. Par ailleurs, depuis le 7 septembre 2022, un 7ème escadrons de gendarmerie mobile est venue renforcer le dispositif opérationnel en Guyane concentrant sur votre seul département un tiers des unités de forces mobiles projeté en outre-mer par ailleurs un renfort judiciaire en provenance de la métropole a accompagné une réorganisation partielle du dispositif sécuritaire, lequel semble porter ses fruits. Lors de la dernière visite de Gérald Darmanin Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, il a pu apprécier l'engagement de l'ensemble des forces de sécurité intérieure coordonné par l'autorité préfectorale. Ainsi, lors des Assises de la sécurité tenue le 30 septembre dernier, il s'est engagé à créer plusieurs brigades dont certaines fluviales ce qui représente 40 effectifs supplémentaires à court terme. Ainsi, il s'est engagé aussi à pérenniser ce 7ème escadron à ce stade, la création de ces nouvelles unités prenant notamment en compte des délais d'interventions liées à l'extension du territoire guyanais est à l'étude et devra prochainement être officialisée. n'en ai pas la date aujourd'hui, mais en tout cas l'engagement est toujours là et le travail est en cours. Monsieur. La parole est maintenant Madame Belletti. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre alors que l'association des maires de France a annoncé en février une hausse de 15% des agressions envers les élus sur un an les données que vous avez rendu public le 15 mars ne sont pas plus encourageantes et des notes au contraire une généralisation de la violence exercée sous toutes ses formes à l'encontre des élus en 2022, 2265 plaintes et signalements contre 1720 en 2021 soit une hausse de 32 101er interlocuteur en particulier dans les petites communes, les maires et les adjoints sont également les premières victimes de cette recrudescence constitue en plus de la moitié des faits recensés en Moselle. Ce phénomène s'est également intensifié ces derniers mois, plusieurs maires ont fait l'objet de menaces d'agressions verbales et physiques. Les élus s'interrogent, ne sachant plus quoi faire face à une agression tiraillés entre leur devoir d'agir pour la commune et la peur omniprésente de représailles pour eux et leurs proches, il pose ouvertement la question aujourd'hui de la poursuite ou de l'abandon de leur mandat. Depuis 2020, 900 maires ont démissionné et le mouvement dans mon département comme ailleurs se poursuit en 2023 à l'aune des violences que connaît actuellement le pays dans sa globalité. La récente loi du 25 janvier 2023, portée par la sénatrice Nathalie Delattre a permis des avancées sur la répression en donnant la possibilité aux associations d'élus au collective unité locale de se porter partie civile afin d'accompagner les élus victimes la principale problématique, à savoir la peur quotidienne dans laquelle vivent les élus locaux restent présentes et pesante. Madame la Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour mettre les citoyens coupables de ces violences face à leurs responsabilités et permettre ainsi aux élus d'exercer leur mandat sereinement. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Rithy je voudrais tout d'abord réaffirmer ma pleine mobilisation avec Gérald Darmanin sur la situation nous apportons notre soutien sans faille à tous les élus victimes d'agressions, chaque jour, la liste s'allonge vous l'avez dit et c'est totalement inacceptable. Je tiens à remercier la police, la gendarmerie et bien évidemment les préfectures qui accompagne les maires dans leur démarche. Comme vous le savez je suis nancéenne mère et je partage le constat que ces atteintes relève avant tout d'une problématique sociétale, lorsqu'un élu est agressé, c'est la République qui est attaqué. C'est aussi toute notre démocratie qui recule. Nous avons chacun pris notre part dans le renforcement de la protection des élus et je remercie comme vous l'avez fait. La sénatrice Delattre qui par sa proposition de loi permet aux associations d'élus, aux collectivités locales au Sénat à l'Assemblée nationale et au Parlement européen de se porter partie civile en cas d'agression d'un élu. J'espère que le Sénat pourra se saisir rapidement d'un texte visant à durcir les peines encourues en cas de violences commises à l'encontre des élus ou de leurs proches. aussi renforcer notre connaissance du phénomène et notre capacité à y répondre pleinement à ce titre avec Gérald Darmanin, nous allons. Créer sans nous avons créé un Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus cette stricte eurent permettra d'avoir une compréhension plus fine du phénomène. Elle devra aussi coordonner la réponse de l'ensemble des acteurs concernés, police, gendarmerie, parquet, préfecture et améliorer la prévention de ce phénomène. Cette annonce est conjointe à plusieurs autres que je ferai dans les prochaines semaines pour recréer la confiance entre les élus et nos concitoyens. J'appelle un choc civique et ce depuis le plus jeune âge, madame la sénatrice dès que ces mesures seront affinées. Je ne manquerai pas de vous rencontrer pour échanger avec vous personnellement sur ce sujet, je vous remercie. Madame belle Haïti. Merci, madame la Ministre, l'exercice d'un mandat local est une grande responsabilité et un grand honneur pour tout citoyen français honneur qui risquent de se raréfier dans les années à venir. Si les élus ne sont pas soutenues à la hauteur de leurs responsabilités. Merci. C'est. Madame Schillinger. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre les zones frontalières sont par nature plus exposés que lire le reste du territoire à la criminalité transfrontalière et à l'immigration illégale. C'est le cas de l'agglomération Ludovic Sienne et plus largement de la zone des trois frontières dans le sud du du département du Haut-Rhin, située à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne et abritant le 5ème aéroport international de France plus de 9 millions de passagers par an. Ce territoire est en effet une des principales portes. De France en terme d'immigration. À titre d'exemple, rien que sur le vecteur ferroviaire franco-suisse, ce sont plus de 5000 migrants clandestins qui ont été interdits. Interpellé par les services français de la police depuis novembre dernier. Dans ce contexte, l'implantation d'un centre de rétention administrative en. De l'euro Airport Mulhouse constituerait une plus-Value certaine dans le soutien à la lutte contre l'immigration illégale et à la mise en oeuvre de la politique migratoire actuellement les centres les plus proches sont situés soit à Geispolsheim soit à Metz Kant, la ville de Saint-, lui, au coeur du territoire des 3 frontières ne disposent-elles que d'un local de rétention administrative de seulement 9 places. Cette situation contraint les agents de police aux frontières à parcourir entre 120 kilomètres et 270 kilomètres pour y accompagner les étrangers en situation irrégulière, les détournant de leur autre mission et accentuant les difficultés qu'ils connaissent déjà du fait que de, du fait du manque d'effectif alors que le gouvernement s'est lancé dans un vaste plan de construction de place de centres de rétention et que le ministère de l'Intérieur a lors de la dernière l'OMPI a réaffirmé sa volonté d'accroître nos capacités de rétention en portant à 3000 l'objectif de nouvelles places, pouvez-vous Madame la Ministre nous indiquer où en sommes-nous de l'art et à Lisa Sion de ce plan et quelles sont les intentions du ministre vis-à-vis du territoire des 3 frontières dont la pression migratoire justifierait qui accueille l'un de ces centres. Je vous remercie. Si Madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Schillinger vous soulignez à juste titre, le besoin de places de rétention dans l'Est qui correspond à un enjeu de premier ordre pour le gouvernement qui porte l'objectif de créer 3000 places en centre de rétention administrative d'ici 2027. Vous l'avez dit. Pour ce faire, une enveloppe de 240 millions d'euros a été votée dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en parallèle une instruction ministérielle du 3 août 2022 a fixé un objectif d'augmentation d'au moins un tiers de la capacité des locaux de rétention administrative Les RA qui permettent de maintenir un étranger en rétention administrative. Vous le savez durant les 48 premières heures

pour l'implantation de nouveau CRA. Il a été décidé de privilégier les projets d'une capacité de 140 places, situé à proximité d'une grande plateforme aéroportuaire, ces projets doivent répondre à la fois un niveau élevé de sécurité bâtimentaire et à une possibilité de démarrage rapide des études et des travaux, ce qui suppose des sites sous maîtrise foncière de l'État ou susceptibles d'être rapidement mis à disposition les projets doivent en outre respecter les contraintes urbanistiques et environnementales. Et permettent la construction d'une salle de justice à proximité immédiate de se sert dans la mesure où les deux CRA existant dans la zone. Elles sont déjà situés dans 2 départements frontaliers de l'Allemagne, la recherche d'un nouveau site paraît devoir privilégier l'objectif d'un rééquilibrage territorial au sein de cette Des propositions seront prochainement formulée par la préfète de la région Grand-Est sur ce point en concertation avec vous-même Merci. Madame Elsa Schalke. au mieux un mandat pour exercer aussi les nombreuses et multiples responsabilité qui incombe désormais est de plus en plus aux maires et aux élus locaux. La question du statut de l'élu local revient régulièrement et on voit bien que l'une des composantes c'est également évidemment la question de la, de la formation, or nous assistons à une baisse notable des demandes de formation, de la part des élus en raison notamment de la complexification de la procédure d'inscription qui exigent depuis octobre 2022, de passer par France Connect, il s'avère que cette sécurisation du dispositif a rendu l'inscription particulièrement complexe, voire même impossible pour les élus locaux. J'ai été alerté en ce sens par l'association des maires du Bas-Rhin en effet des élus ont pu rencontrer de très nombreuses difficultés pour créer une nouvelle identité numérique pour attester de l'identité ou encore avec des problèmes de validation des données saisies. Madame la Ministre toutes ces démarches décourage davantage qu'elles encouragent ce qui est profondément effectivement dommageable notamment pour l'exercice. Du mandat et à l'heure où nous décompte ont malheureusement près de 4000 et élus démissionnaires en trois ans dont près de 1000 maires à quel point l'exercice des responsabilités locales est devenue difficile, délicat mais ô combien précieux pour la vie de nos communes. Il est nécessaire que ces dispositifs soient simple clair pragmatique et utilisable et j'aurais rappellerai que les élus locaux cotisent. À hauteur de 1% pour financer ce droit individuel à la formation d'où ma question, madame la Ministre, qui est très simple, comment comptez-vous faire pour améliorer ce dispositif et le rendre le plus simple c'est une attente très forte de la part des élus locaux. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Schalke depuis janvier 2022, les élus peuvent directement mobilisés leur droit individuel à la formation via mon compte élu une plateforme numérique adossé à mon compte formation, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et des consignations, vous le savez. Face aux nombreuses fraudes sur la plateforme. Le gouvernement a mis en place des mesures de sécurité renforcées afin de préserver les droits des utilisateurs. Le niveau supérieur de sécurité, de France Connect appeler France Connect plus est déployée depuis le 25 octobre 2022 pour l'achat d'une formation sur mon compte formation et mon compte élu pour ne pas dissuader les personnes souhaitant s'engager dans une démarche de formation. Un dispositif complet d'accompagnement, été mis en place par la Caisse des dépôts et des consignations et par la poste adapté en fonction des besoins identifiés parmi lesquels évidemment ceux des élus locaux, une communication large, comprenant des informations pratiques et des tutoriels a été diffusée auprès des acteurs concernés, cela reste difficile, j'en suis consciente. Si, en dépit de ces outils des usagers rencontrent des difficultés pour générer leur identité numérique. Il faut qu'ils se rendent dans les bureaux de poste, il faut qu'il se rende, il faut qu'ils se fassent accompagner par des conseillers numériques c'est vrai enfin une assistance téléphonique dédiée aux élus locaux a été mis en place un numéro spécifique leur permet de contacter un interlocuteur pour répondre à leurs questions. Le gouvernement tiendra compte des difficultés engendrées par ces évolutions récentes du temps nécessaire à l'appropriation par les élus de cette nouvelle procédure après concertation avec les associations d'élus, il a été décidé de relever de 700 euros à 800 euros le plafond des droits pouvant être détenues afin de ne pas pénaliser les élus qui n'ont pas utilisé leur droit en 2022 et qui bénéficieront ainsi en 2023, 2023 pardon d'un abondement de 400 euros, portant le montant total de leur compte formation à 800 euros. Ceci étant, le travail se poursuit et l'amélioration doit être réalité pour encourager la formation de nos élus. Vous avez tout à fait raison. Merci madame Challes quelques secondes. Je vous remercie effectivement Madame la Ministre c'était important de relever le plafond mais il est. Précieux que justement en fait l'ensemble des difficultés soit levée pour éviter en fait tous les freins et toutes les difficultés que les élus locaux nous relaye systématiquement et quotidiennement, je vous remets. Si la parole est à Pierre lourd. Madame la ministre ma question porte sur les conséquences de la compensation de la CVAE notamment mais plus généralement sur la baisse des la suppression des impôts locaux au bénéfice d'une fraction de TVA. La CVAE et la baisse des impôts de production de l'État a mis en place la compensation des fraction de TVA. Néanmoins, il apparaît que ce changement de mode de financement. N'est pas aussi optimale que souhaité. Tout d'abord la TVA a pris au fil des années une part de plus en plus importante dans les Budgets des collectivités et cela s'est fait au détriment de l'État qui en 2021 ne percevait plus que la moitié de ses recettes totales. Par ailleurs la CVAE dépendait auparavant de l'activité des territoires à un moment où on veut faire revenir des entreprises industrielles sur nos territoires, y compris sur les territoires ruraux. Il n'y aura plus beaucoup d'intérêt pour les collectivités d'investir. Dans. Ses perspectives. Dans ce contexte économique déjà difficile une compensation à l'euro près de la CVAE qui tarde à venir. Deuxièmement, la suppression de ses impôts locaux à diminuer drastiquement l'automne diminue drastiquement Cette réforme a donc créé une rupture entre fiscalité et territoires. Ce qui amène la Cour des comptes en octobre 2022, a évoqué une nouvelle proposition de réforme pour recentrer la fiscalité locale sur le bloc communal. En accord avec les objectifs d'autonomie financière des collectivités. Il lui demande quelles sont les réflexions et les pistes actuelles, autour de cette réforme. Madame la ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le Sénateur lourd. Comme vous le savez. Afin d'accroître le pouvoir d'achat des ménages afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, le gouvernement a souhaité supprimer la taxe d'habitation sur les résidences principales, pour l'ensemble des foyers fiscaux ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises la CV les communes ne perçoivent donc plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Depuis 2021, mais elle bénéficie en contrepartie du transfert de la taxe foncière des départements. Ce transfert a permis de préserver leur pouvoir de taux sur un montant identique à celui perçu auparavant au titre de la taxe d'habitation. Les EPCI à fiscalité propre et les départs. Autrement perçu en contrepartie de leur perte de taxe d'habitation, de taxes foncières une fraction de TVA très dynamique. Celle-ci a progressé de plus de 902.022 et devraient progresser de 6% en 2023, la part régionale de la CVAE a été supprimé en 2021, les régions perçu en contrepartie une fraction dynamique de la TVA à hauteur de leur montant de CVAE perçue en 2021 cette compensation est d'autant plus favorable aux régions que la TVA a progressé de plus de 9% en 2022. La suppression de la part de CVAE du bloc communal et des départements a fait l'objet d'une compensation par l'intermédiaire d'une fraction de TVA toujours dynamique pour tenir contre de la dynamique spécifiques à chaque territoire, la dynamique de TVA, affectée au bloc communal, abonde un fonds national dont un décret d'application fixera les critères de répartition très. Bientôt. Au total, c'est plus de 50 milliards de TVA qui sont versés aux collectivités territoriales en 2023 ils traduisent une compensation intégrale pérenne et dynamique de la suppression à la fois de la taxe d'habitation et de la CVAE. Mais je pense que vous saviez tout ça et en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. Si Monsieur. Oui, madame la ministre, effectivement c'est tout cela. On dit aussi, on lit aussi que la situation financière des collectivités territoriales s'est améliorée c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour les départements, c'est beaucoup moins vrai pour les communes et les collectivités très local et puis on perd ce lien avec les citoyens. Chaque service à un coût et finalement aujourd'hui ben il suffit de réclamer ça n'a plus de coups. Personne ne sait d'où vient l'argent alors que quand on touche le portefeuille. De ses les Lecteurs de sa communauté, hé bien là il y a un relais Direct entre le citoyen et les élus locaux. merci. Madame la présidente Billon. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre afin de pouvoir bénéficier de la réfraction de la TGAP votre ministère à imposer l'installation d'un compteur homologué avant le 31 décembre 2022. Si l'homologation du compteur de la Marsick date de 2018. L'homologation d'un second compteur de marque Fuji date de novembre 2022. Vous n'ignorez pas que nombre d'opérateurs utilisent le compteur de Marc et Merson reconnu fiable et permettant de bénéficier de la réfraction de la TGAP jusqu'à ce jour ça notamment le cas du syndicat vendéen de traitement de déchets, tu Rivalis. Or, pour des raisons que nous ignorons le compteur Emerson n'est pas homologué et obligations et de notre fête aux opérant aux opérateurs d'investir dans un système homologué pour continuer à bénéficier de cette réfaction avec la mise en concurrence seulement rendu possible de novembre 2002. En novembre 2022, le temps des procédures administratives et la durée des travaux ne permettent pas l'installation de nouveaux compteurs avant le 2ème semestre 2023 en conséquence les opérateurs pourraient être De plus, cela semble peu pertinent d'imposer à des collectivités d'acquérir un nouvel équipement, alors que la réfaction de la TGAP ne sera plus possible au 1er janvier 2025, soit dans moins de 2 ans. C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise des investissements et compte tenu des délais contraints, pour les procédures administratives, je vous demande s'il peut être envisagé que les compteurs de Marc Emerson soit maintenu pour bénéficier de cette réfaction de TGAP merci. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Billon vous interroger le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires Christophe Béchu sur l'obligation pour les exploitants de décharges de disposer de compteur de biogaz homologué pour pouvoir bénéficier d'un tarif réduit sur la taxe générale sur les activités polluantes ne pouvant être présent il m'a chargé de vous répondre. Il existe en effet un tarif réduit sur cette taxe lorsque l'installation valorisent le biogaz capter le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et conscient des difficultés. Passées d'homologation. C'est pourquoi, avec le ministère en charge du Budget nous avons repoussé à plusieurs reprises l'entrée en vigueur de cette condition pour accéder au tarif réduit. Initialement prévue pour le 1er janvier 2020, celle-ci est entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Néanmoins, nous entendons vos arguments et les difficultés auxquelles les opérateurs font face. C'est pourquoi nous tenons à vous informer que nous avons prévu de reporter à nouveau l'entrée en vigueur de cette obligation au 1er janvier 2024. Ce report sera officialisée par un arrêté que nous allons publier conjointement avec le ministère en charge du budget dans les prochaines semaines, la valorisation du biogaz des décharges fait aujourd'hui partie des solutions pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et contribuer à notre souveraineté énergétique le tarif réduit de taxation en prend acte. Je rappelle toutefois que cette réduction n'a pas vocation à durer la généralisation du tri à la source des déchets alimentaires et des déchets verts à compter du 1er janvier 2024 prévu par la loi anti-gaspillage de 2020 et par le droit européen conduira en effet à une montée en puissance de solutions de valorisation de ces déchets fermentescibles plus efficace. Comme le compostage ou la méthanisation. Je vous remercie. merci monsieur le président. Merci madame la ministre. Alors nouveau délai 2024 OK sauf qu'a priori la réfaction de la TGAP ne sera plus possible en au au 1er janvier 2025, donc à défaut de, de progrès de de reporter encore la réfaction et le l'impossibilité de le faire, je, je me dis qu'il aurait été préférable de pu avoir de délai du, du tout, puisque finalement. On demande des investissements supplémentaires donc on alourdit les finances publiques. J'aurais souhaité que finalement les délais soient supprimés. Je vous remercie, madame la ministre. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de communes a été acté par la loi dite notre le Sénat s'est opposé à cette réforme car il était conscient des difficultés qu'il allait se poser pour les communes rurales. Le Sénat a tenté d'obtenir le rétablissement du caractère facultatif de ce transfert à de nombreuses reprises lors d'examen de cinq textes pas moins différents. En janvier 2017 avec la loi dite Retailleau voté à l'unanimité en octobre 2007, les députés ont renvoyé ce texte en commission. En décembre 2019 avec la loi dite engagement de proximité. La commission mixte paritaire n'a pas été conclusive sur ce point, la loi dit tout 3DS n'a pas permis d'avancer sur cette question. Ensuite des assouplissements ont été obtenus avec le report au 1er janvier 2026 de ce transfert et le maintien des syndicats infra-communautaire après cette date. Le 16 mars de cette année. Le Sénat à revoter à une large majorité. La. Le caractère facultatif de ce transfert. Et donc je ma question c'est, je souhaite savoir si cette petite loi sera mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et quand.

d'exercice des compétences eau, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines. L'article L 52 14 tiré 16 du code général des collectivités territoriales a ainsi institué un mécanisme de délégation de ses compétences et dispose de cette délégation au profit d'un syndicat mentionnés à l'article L. 52 12 tirer hein existant au 1er janvier 2019 et inclut en totalité dans le périmètre de la communauté de commune. C'est important de rappeler ces assouplissements même si je suis très au fait de ce qui s'est passé au Sénat il y a pas si longtemps que ça, puisque j'étais au banc pour ces territoires ayant utilisé ces possibilités, le mécanisme est perçue comme un moyen de maintenir des structures historiques dotée de moyens techniques et humains adaptés ou comme un moyen d'assurer la continuité du service, le temps que le PCI soit en capacité de reprendre la compétence, lors de la présentation du plan eau par le président de la République et par Christophe Béchu Ministre de la Transition écologique et de la coopération des territoires de la cohésion des territoires, il a été rappelé le besoin essentiel de la mutualisation pour la protection de nos ressources en eau besoins essentiels de la mutualisation cette mutualisation sera prochainement étudiée par une mission parlementaire au Sénat. Il a été rappelé que le président de la République ne souhaitait pas revenir sur l'obligation de transfert. Contrairement à ce que la PPL elle a voté au Sénat mais qu'il souhaitait l'intégration d'une logique de différenciation ce dialogue qui s'engage avec le Sénat est pour moi essentiel dans cette trajectoire vital de préservation de la ressource en eau et pour son acceptation par l'ensemble des élus locaux. Je vous remercie. Oui, madame la ministre, je vous remercie. Je sais qu'il y avait eu des assouplissements, mais vous savez comme moi qu'il ne conviennent pas du tout parce que finalement le prix unique, de l'eau dans la communauté de communes et subsiste et il y a des communes qui vont voir leur leur prix augmenter. Alors qu'il y a il il y a rien de nouveau et donc ça ne convient pas et je vous fais une proposition, on sait qu'on va qu'on va manquer d'eau qu'on aurait des difficultés parce que le climat change et par conséquent il faut trouver des solutions. Il existe dans certains départements, des syndicats départementaux de production d'eau et de transport d'eau et moi je vous propose le faire une, un projet de loi, en disant que dans les départements où il y en a pas, hé bien les départements doivent faire un syndicat départemental d'eau pour la production et le transport d'eau à charge pour les communes de de de la distribuer et ça règle. Après la question, merci aussi d'eau. Merci de cette proposition et la parole est à monsieur Cyrille va. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi climat adoptée en 2021 est venu interdire l'utilisation de chauffages extérieurs dans l'espace public. Cette interdiction est officiellement entré en vigueur en mars 2022, date de la publication du décret d'application de cette mesure. Si c'est si avait comme objectif principal d'interdire les chauffages extérieurs en terrasse. La question des commerces non sédentaires semble avoir été occulté des commerçants itinérants ont en effet besoin de pouvoir se chauffer lorsqu'ils exercent leurs activités en extérieur durant l'hiver par exemple sur les marchés. Les températures sont souvent négatives durant cette période, l'utilisation d'un chauffage d'appoint est donc indispensable pour qu'ils puissent exercer dans de bonnes conditions. Or puisqu'aucune dérogation à l'interdiction n'est prévue par le décret pour ce cas de figure, de nombreux commerçants indique qu'il est désormais courant que la police municipale leur demandent de couper leur chauffage ou les contraventions. Cette interdiction d'utiliser un chauffage d'appoint et dangereuse à la fois pour la santé de ces commerçants. Certains en faisant état d'engelures ou de problèmes de circulation sanguine. Et pour avoir été fils de maraîchers en fait les marchés pendant une trentaine d'années, je peux vous assurer que c'est pas un mythe. Il y a aussi un impact sur les produits et notamment les denrées périssables et aussi un impact sur la leur activité puisque dans ces conditions il ne aurait pas possible d'exercer des 12 mois pleins. Une telle baisse d'activité pour grandement atteinte à la vitalité de les territoires ruraux dans lesquels les commerces itinérants sont essentielles pour l'accès à de nombreux produits et denrées les territoires de montagne sont les plus impactées puisqu'ils enregistrent des températures les plus extrêmes aussi Madame la Ministre je souhaiterais savoir si vous comptez prévoit une dérogation c'était interdiction des systèmes de chauffage dans l'espace public en faveur des commerçants non sédentaires. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Pell va à la Convention citoyenne pour le climat a proposé une action globale de réduction de la consommation d'énergie dans les espaces publics et bâtiment tertiaire concernant le chauffage, l'éclairage et la climatisation. Elle a recommandé l'interdiction de chauffer les espaces publics extérieurs sur ce gaspillage d'énergie. Le législateur a repris cette proposition à l'article 181 de la loi. Numéro 2021 tiré. 11 04 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets en vertu du nouvel article L 21 du code général de la propriété des personnes publiques l'utilisation sur le domaine public de système de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. Cette disposition un Champ large le législateur a posé une interdiction générale des espaces extérieurs chauffés ou climatisés couvrant tout le domaine public sans distinguer l'activité concernée. Le décret 20 22 tiré 452 du 30 mars 2022 pris pour l'application de cette disposition législative a uniquement exemptés de l'interdiction les lieux couverts et fermés de manière étanche à l'air et les installations mobiles couverte et fermée nécessaires à l'animation de la vie locale qu'il s'agisse des activités foraines circassienne des manifestations culturelles, sportives, festives culturelles ou politiques. Par conséquent, les activités qui se déroule sur le domaine public à l'air libre tels que l'activité de commerces ambulants sont soumises à cette interdiction de chauffage extérieur nous en comprenons les les effets cependant. on précise que le chiffre d'affaires des commerçants en extérieur ne devrait pas être trop impacter car cette interdiction ne vise pas l'énergie nécessaire à la production ou à la conservation des denrées vendues elle ne pénalise que les clients qui doivent se couvrir un peu plus. Je vous remercie.

on est quand on doit mettre on passe les bâches qui sont gelés. On ne peut pas le faire avec des gants derrière on a des légumes à l'intérieur aussi qui sont des denrées périssables qui s'abîme donc. Donc l'impact il est plutôt global et ça, je parle sur toute une thématique. Donc il serait bien de pouvoir quand même une une mesure dérogatoire spécifique pour. Ses. Domaines d'activité, notamment sur les sur les marchés. Je leur ai dit surtout sur des territoires de montagne comme les nôtres où les températures sont négatives et ça sur trois ou quatre mois de l'année. Je vous remercie. Merci Monsieur le Rudulier. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre le loup est dans la bergerie et plus précisément aux portes de Marseille depuis des années le loup avance pas à pas sur le territoire provençal jusqu'à élire domicile dans le massif des Calanques aux abords donc de l'agglomération marseillaise, le 1er mal a été repéré il y a à peu près 2 ans dans le massif de Saint-Cyr depuis pas moins d'un couple cinq louveteaux et un mâle adulte ont élu domicile dans le parc des calanques. Les éleveurs, les agriculteurs connaissent bien les dangers liés à la présence du loup autour de leurs pâturages et surtout de leurs élevages. L'agriculture extensive et le pastoralisme sont des traditions ancestrales et une part fondamentale de notre Patrimoine immatériel de notre région mais ses traditions et c'est Patrick sont aujourd'hui mises en péril par le retour du loup. Avec notamment un déséquilibre des espaces naturels. Il est donc impératif que les pouvoirs publics puissent revoir les mesures d'accompagnement, notamment les dispositifs d'aide à la protection des des troupeaux et les procédures d'indemnisation filer gardiennage chiens de protection. Tirs d'effarouchement prélèvements encadré des solutions existent alors Madame la Ministre comment comptez-vous défendre le pastoralisme. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Le Rudulier. L'action du gouvernement concernant le loup vise à concilier les activités d'élevage et la préservation de l'espèce, strictement protégée par le droit national, européen et international. Le loup peut toutefois occasionner des dommages sur les troupeaux pour soutenir l'élevage et lutter contre la prédation le plan national d'action 2018 2023 sur le loup et les activités d'élevage permet entre autres le financement de moyens de protection des troupeaux et l'indemnisation des éleveurs. Le préfet des Bouches-du-Rhône a par arrêté du 31 juillet 2023. Pardon. 31 janvier 2023 délimiter les zones d'éligibilité du département à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation par le loup pour l'année 2023, classement des communes encercle un, deux ou trois selon le risque ou l'intensité de prédation permet aux éleveurs d'ovins et de caprins de répondre à l'appel à projet national visant à les accompagner financièrement à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en compensant les surcoûts induits. Par les changements de pratiques un travail de revalorisation des montants d'indemnisation des coûts directs des attaques est en cours. Comprenant les animaux morts ou qui ont nécessité une euthanasie et les animaux disparus non tenues en parc clos est également en cours. Une étude visant à recalculer le coût des pertes dire dites indirectes consécutive à la perturbation du troupeau, du fait notamment du stress de la moindre prise de poids des avortements de la baisse. De lactation, conformément à la législation et en plus de ce que je viens de vous dire et de ses travaux en cours. Conformément à la législation communautaire et national des dérogations à la protection stricte du loup peuvent être utilisées, elles permettent d'autoriser des tirs de loups dans la limite d'un plafond fixé chaque année de matière à respecter la viabilité de la population. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre défendent le le pastoralisme c'est également défendent les centaines d'éleveurs, agriculteurs qui défendent nos traditions mais qui contribuent à à nourrir de manière très qualitative, les bucco-rhodaniens mais également des millions de Français, mon propos n'était pas l'éradication du loup puisque c'est une une espèce protégée par la la convention de Genève de 1979. Mais c'est bel et bien de de garantir aux agriculteurs, aux éleveurs, la pérennisation de de leur activité, les pouvoirs publics leur dois bien ça je pense. Merci beaucoup. Si Madame Loisier. Merci monsieur le président, madame le Ministre, mes chers collègues. Moi, je souhaite attirer votre attention sur la mise en oeuvre d'une loi qui nous est cher au Sénat, c'est la loi, Didier de 2014 qui vise à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art je de rétablissement des voix c'est tout. Ce sont donc les ponts construits en l'occurrence pour établir une voie de communication appartenant à une collectivité interrompue par une infrastructure de transport de l'État ou les établissements publics. On pense bien sûr à VNF. À la SNCF ou réseau routier ferroviaire et fluvial. Afin de faciliter la gestion de ses ouvrages et et le coup et prévenir leur détérioration cette loi d'initiative sénatoriale, donc de 2014 a prévu que ces ouvrages feraient l'objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voix et franchi ces conventions devait préciser le rôle de chacun. Quant à la gestion des ouvrages au niveau opérationnel, c'est-à-dire les modalités d'intervention mais également les modalités de répartition du financement entre les différents propriétaire ou gestionnaire des voies relatif donc à la surveillance à l'entretien à la réparation renouvellement donc des conventions absolument essentiel. Un recensement un recensement été publié en juillet 2020 en Côte-d Or et qu'il a, il a permis d'identifier les ponts soumis à cette loi. La plupart aujourd'hui se dégradent et présente de nombreux problèmes de sécurité, de circulation et les collectivités locales restent dans l'attente de ces conventions afin d'engager légalement les travaux selon les maires et les élus locaux qui sollicitent Voies navigables de France, l'établissement de la convention de répartition des charges reste aujourd'hui suspendu sans aucun argument tangible ce retard à organiser l'organisation publique conformément à l'esprit de la loi et donc préjudice préjudiciable aux usagers mais elle expose aussi les collectivités, les maires à une insécurité à la fois juridiques et financières et aujourd'hui, ils ne peuvent plus attendre. Madame la Ministre je souhaiterais donc savoir si les élus doivent solliciter en urgence la médiation du préfet prévue dans l'instruction du gouvernement du 15 mars 2018 pour activer ce dossier et d'autre part pourquoi les ponts soumis à la loi et donc à convention ne seraient pas éligibles au programme national pont comme l'indiquerait aujourd'hui le CEREMA aux élus. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci monsieur le président, madame Ana sénatrice loisirs donc comme vous l'avez rappelé la loi 2014 tirer 774 du 7 juillet 2014, dite la loi Didier. A pour objet de répartir par convention les charges financières relatives à la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement des ouvrages d'art de rétablissement des voix interrompue par une infrastructure de transport entre d'une part les propriétaires ou les gestionnaires des voix portée et d'autre part ceux des voix franchi. Elle ne remet pas en cause la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle ces ponts sont des éléments constitutifs des voix dont ils assurent la continuité par conséquent les collectivités de me responsable de leurs ouvrages. Elles sont tenus de réaliser tous les travaux nécessaires pour empêcher leur dégradation et assurer leur sécurité. La contribution du gestionnaire de la voix franchi et de nature financière. La maîtrise d'ouvrage ne lui étant pas transférer concernant plus particulièrement Voies navigables de France qui a la responsabilité de 6700 kilomètres de réseau, la prise en charge de ces coûts ne peut être que progressive en raison du grand nombre d'ouvrages ah conventionné et du temps nécessaire pour rassembler des bonnes connaissances techniques pour une grande partie de ceux-ci. Si la négociation comme vous l'avez indiqué pour conclure une convention de répartition n'a pu aboutir. Alors la loi Didier prévoit en effet une médiation du préfet du département, à la demande d'une des parties. Enfin, concernant le programme national pont il n'a pas le même objet. Il vise à aider de petites communes pour la gestion de leurs ouvrages et non à financer des obligations incombant à l'État ou à ses opérateurs au titre de la loi. Il n'a donc pas vocation à traiter ces ouvrages de rétablissement sauf entamer une ressource précieuse pour les communes. Je vous remercie. Oui. Merci monsieur le président, madame la ministre, s'il constitue une incitation accrue à la rénovation énergétique et constitue à ce titre une dimension louable par rapport à l'ancien dispositif. Le dispositif de le diagnostic pardon de performance énergétique n'en demeure pas moins en l'état problématique dans sa mise en application concernant le bâti ancien les territoires. Et je pense là Madame la Ministre notamment au petit Patrimoine, non protégé souvent. Et à sa préservation. De nombreux dysfonctionnements été mises en lumière soit dans les outils de calcul des diagnostiqueurs soit dans la formation et sa mise en oeuvre est l'objet de nombreuses contestations et difficultés de fait mode et méthodes de construction contemporaine standardisées inadaptées s'avère dangereuse pour la préservation des bâtiments anciens. Cette situation est particulièrement préjudiciable et met en péril le Patrimoine local véritable vecteur d'attractivité des territoires. J'attire d'ailleurs votre attention sur les comptes. Les conclusions de la table ronde organisée le 1er février dernier par la Commission de la culture de l'éducation et de la communication du Sénat consacrée à la transition écologique du bâti ancien qui a permis de rappeler que la rénovation de l'existant était à privilégier plutôt que de s'orienter vers la construction neuve, tout en concluant à la nécessité d'adapter la réglementation aux spécificités du du Patrimoine vernaculaire. Dès lors, comment comptez-vous faire évoluer le DPE et ces critères. Quant aux caractéristiques du bâti ancien, véritable Patrimoine local et selon quelle méthodologie. Cela nécessite également d'outiller les professionnels pour y répondre et comment peut-on envisager ce point. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, de Nicolas il la rénovation des bâtiments existants constitue une priorité pour notre gouvernement. Le diagnostic de performance énergétique le DPE un outil central dans cette politique de rénovation. La réforme de 2021 a permis de fiabiliser le des. En rendant plus fiable sa méthode de calcul et s'est donné d'entrée s'agissant du bâti ancien qu'on vient de rappeler qu'aucune réglementation thermique s'appliquant à la construction neuve n'existait avant 74. On ne peut donc aujourd'hui. Avoir aucune certitude sur le niveau de la performance énergétique des bâtiments construits avant 1974 en se basant seulement sur leur année de construction cette réalité se traduit dans la méthode du DPE par la définition de valeurs par défaut différencié en fonction de l'année de construction avec donc des valeurs par défaut moins bonne, le recours à ces valeurs par défaut doit toutefois être éviter autant que possible afin de définir plus précisément la performance énergétique d'un logement. Par ailleurs, la réforme de 2021 sur le DPE a permis de mieux considérer certaines spécificités de certains bâtiments anciens, la nouvelle méthode du DPE tient compte de la forte inertie de certains matériaux présents dans le bâti ancien terre Pierre briques ancienne colombage en adaptant sur certains mois de l'année les besoins de chauffage et de refroidissement au regard de ce qui précède, aucune évolution de la méthode du DPE pour le bâti ancien n'est envisagée à court terme. Néanmoins, il y a un enjeu. Sur la qualité de la réalisation des DPE. Le ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein a annoncé récemment le renforcement à venir de la formation et des contrôles des diagnostiqueurs DPE. Enfin le gouvernement soutient l'expérimentation d'un Label de performance énergétique pour la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Je vous remercie. Merci monsieur le président, madame la ministre. Alors que la gestion de l'eau, des frais. L'actualité, permettez-moi d'évoquer un problème qui touche à nappe phréatique d'Alsace qui est la plus grande ressource en eau en Europe dans les années 50, l'État a construit un canal long de 50 km par aller. Utilisés pour la navigation et pour l'hydroélectricité ce canal étanche empêche l'alimentation par infiltration naturel de la nappe phréatique, avec un volume manquant chiffré à un milliard de mètres cubes par an. Les conséquences en ont été un abaissement de plusieurs maîtres de la nappe un assèchement des puits des rivières et des zones humides. Pour limiter les effets de ces aménagements et suite à des manifestations. L'État a construit un canal d'irrigation en béton alimentés grâce à des droits d'eau sur le Rhin qui permettent une recharge de la nappe de plus de 500 millions de m3 par an. Mais depuis une vingtaine d'années, l'État laisse ce réseau tomber en ruine réduit son alimentation au tiers de sa capacité quand ils ne le coupe pas à certaines saisons. Les effets désastreux de cette politique se feront sentir par des périodes de stress de la nappe phréatique de plus en plus fréquentes et des rivières à sec. Le syndicat j'aime à bien des canaux et rivières de la Plaine à solliciter l'état à plusieurs reprises pour qu'on lui transfère ses ouvrages et que vous fassiez appliquer les contrats de concessions hydroélectriques du Rhin qui stipule que l'énergéticien doit prendre à sa charge les frais liés à son impact sur la nappe. Ce syndicat souhaite transformer ses canaux bétonné en rivière naturelle pour développer la biodiversité ré-alimenter la nappe par infiltration naturelle. Malheureusement, l'État fait la sourde oreille. Ma question est donc simple, quand est-ce que l'État acceptera de s'asseoir à la table des négociations avec le syndicat. J'ai ma pierre du secteur et s'engagera à faire respecter la loi et les conditions de contrat de concession. Merci. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Draxler au sein de l'État, c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire le Masa et non le ministère de la transition écologique et des collectivités territoriales qui est actuellement propriétaire des canaux d'irrigation de la harpe qui sont en pratique géré par la Direction départementale des territoires du Haut-Rhin. Ces canaux ne sont pas bétonné et donc ne sont pas étanches sur toute leur longueur il réalimente la nappe. Grâce aux droits d'eau agricole. Ils sont entretenus par l'État pour rester fonctionnel et reste dans un état que nous jugeons convenable. Ils permettent un transite d'eau avec un début, un débit toujours maintenu et même sur une plus longue période. Le chômage divers ayant été nettement réduit. L'État est favorable à un transfert vers une collectivité territoriale et la exprimé depuis de nombreuses années une collectivité pourrait mener un ambitieux projet de renaturation en allant au-delà des besoins agricoles strict. Des discussions ont été menées par le Masa avec le département du Haut-Rhin, puis avec la collectivité européenne d'Alsace depuis la création de celle-ci. Une stratégie de transfert est en cours d'élaboration par le Masa en collaboration avec les services déconcentrés de l'État concerné. Celle-ci doit permettre d'assurer la transmission du foncier des ouvrages et des moyens humains et financiers dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Mais Madame la Ministre, nous avons un syndicat local qui est vraiment motivés et volontaires pour travailler sur ce dossier. Je crois qu'il faudrait peut-être leur donner l'occasion aussi de vous faire part de, de cette volonté. Merci beaucoup. Merci. Dernière question pour cette séance. Madame Ract-Madoux. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre en 2019, la refonte de l'offre du RER D. Sur l'ensemble de la région capitale devait résoudre les retards sur la ligne et améliorer le confort pour les 615.000 usagers quotidiens de la ligne. En réalité les dysfonctionnements n'ont pas cessé. Et la solution technique adoptée oblige désormais de nombreux usagers des branches sud à une rupture de charge, c'est-à-dire à changer de train en gare de Corbeil ou de Juvisy et entraîne un allongement du temps de parcours de minimum 15 minutes par trajet. Je souhaite saluer l'initiative des élus de 6 communes de la ligne Bâle-. Corbeil-Essonnes étiole Malesherbes Ris-Orangis et Soisy-sur-Seine et les associations d'usagers de la ligne dure. Qui ont ensemble missionné un bureau d'études suisse indépendant pour chercher une solution alternative et crédible. Cette étude a montré que la création d'une nouvelle ligne, l'AS pourrait permettre dès 2025 de diminuer le temps de parcours de près de 18 minutes sur le tronçon Corbeil-Essonnes Gare de Lyon et sans correspondance. IDFM a confirmé que cette étude serait bien pris en compte dans le cadre de la révision du schéma directeur du RER D. Tout en précisant que des études complémentaires sont nécessaires. De leur côté les élus viennent déjà de commander un complément d'étude pour affiner certains points notamment la question du matériel. Cette création pourrait améliorer significativement et à un coût raisonnable, la vie des usagers de ce transport du quotidien. Aussi au regard des engagements pris par la Première ministre. Le plan d'avenir pour les transports et la reprise des négociations sur le volet mobilité du CPER en Île de France, je vous demande Madame la Ministre, comment le gouvernement peut apporter son soutien à nos transports du quotidien et à la prise en compte de cette ligne s et son intégration dans le cadre de la révision du schéma directeur du RER D pour une étude en 2023 et un test en 2024. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Ract-Madoux. Comme vous le savez, l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France relève de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité Île-de-France mobilités IDFM l'État mobilisés aux côtés de la région pour investir dans les infrastructures de transport ne peut toutefois pas se substituer aux collectivités ou leurs groupements sans contrevenir au principe de libre administration des collectivités locales les conclusions de l'étude du bureau d'études suisse SMA sur la faisabilité d'une ligne. De RER, reliant. Malesherbes Melun à Paris. Avec des missions directes entre Juvisy et Paris réalisé à la demande d'élus des communes concernées permettront effectivement d'éclairer les suites qu'IDFM compte donner à ce projet. Elles pourront être discutés dans la concertation en cours pour la révision du schéma directeur de la ligne du RER D, à laquelle les associations d'usagers et les maires des communes concernées participent. Pour ce qui le concerne à l'État soutient le développement des réseaux de transport collectif via les contrats de plan État-Région, comme vous l'avez dit, comme cela a été le cas avec le CPER 2015 2022, une enveloppe importante sera mobilisée par l'État pour le réseau RER sur la nouvelle contractualisation 2023 2027 dont les négociations avec les collectivités menée par le préfet de région débuteront très prochainement. Ces négociations permettront d'aborder l'intégration du financement d'une éventuelle création de cette ligne-ce au regard notamment des conclusions des études complémentaires en cours et d'arbitrer le plan de financement du projet dit du terrier de Bercy qui permettrait d'accroître à plus long terme, au-delà de 2032 les capacités d'insertion de train une vigilance toute particulière devrait être conservé puisque sur l'axe cohabitent également des trains de longue distance vers Clermont-Ferrand par exemple je vous remercie. Très bien je vais suspendre la séance. Merci madame la ministre, elle sera reprise à 14h 30 pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant fusion des filières responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier la séance.